d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,

Monsieur le Premier ministre, le variant delta ouvre un nouvel épisode de l'épidémie de covid, qui, une fois de plus, prend le monde entier à contre-pied. Les pays d'Asie et du Pacifique qui ont adopté la stratégie du « zéro covid » et n'ont pas centré leurs efforts sur le vaccin font face aujourd'hui à de nouvelles flambées. Les pays pourvus de vaccins chinois et russes, distribués pour des raisons de propagande, sans les contrôles nécessaires, s'aperçoivent qu'ils ne protègent pas et sont aujourd'hui massivement touchés. Quant à l'Europe, moquée au début de l'année pour son retard et sa prudence, on peut se réjouir qu'elle dispose aujourd'hui des vaccins les plus efficaces. Malgré les campagnes des complotistes et des « antivax », ses populations sont désormais les plus vaccinées derrière celles des États-Unis et d'Israël. Enfin, à partir du 1 juillet, elle sera le principal producteur et distributeur de vaccins pour le monde entier. Cependant, la course de vitesse entre l'immunisation de masse et la dissémination du virus, qui semblait en bonne voie d'être gagnée, est remise en cause par le nouveau variant, plus contagieux, et la vaccination commence à marquer le pas. Le risque est clair : celui d'une quatrième vague à l'automne. Particulièrement préoccupant est le taux de vaccination des personnels de santé- pour certaines catégories, il n'atteint que 50 % ! -, mettant ainsi en danger ceux qu'ils sont censés soigner. Beaucoup de scientifiques conseillent la vaccination obligatoire, au moins dans certaines professions et pour les publics à risque, à l'instar d'autres vaccins pour les soignants. Devant cette nouvelle escalade du risque, ne pensez-vous pas qu'il va falloir envisager des décisions en ce sens avant l'automne ?

Nous sommes tous attachés à la liberté individuelle, mais lorsqu'elle est invoquée par ceux qui refusent le vaccin, elle équivaut, en fait, à la liberté de mettre en danger la vie d'autrui. Il s'agit non plus de liberté, mais d'égoïsme

qui est déjà à l'oeuvre dans de très nombreux pays du monde, pas toujours très loin de la France. Vous l'avez rappelé, il est extrêmement contagieux, beaucoup plus que les variants qui l'ont précédé. Point très positif,

notre propre situation sanitaire. Apparemment, mesdames, messieurs les sénateurs, grâce aux efforts collectifs des Françaises et des Français, ainsi que de toutes les collectivités publiques, notre situation est orientée très favorablement. Vous connaissez toutes et tous la situation du taux d'incidence, les baisses très fortes du nombre de malades hospitalisés, dans les services de réanimation en particulier, le nombre de décès, etc. Pour autant, vous avez parfaitement raison, il est de notre devoir d'anticiper les évolutions que l'on constate partout en dehors de chez nous. Nous avons très largement commencé de le faire.

même si- j'en profite pour en informer le Sénat -, ces derniers jours, les prises de rendez-vous sont reparties à un rythme beaucoup plus satisfaisant. Je parle bien entendu des prises de rendez-vous pour les primo-vaccinations, la seconde injection marchant bien.

de l'Assemblée nationale et du Sénat pour savoir quelles sont leurs propositions sur tous ces sujets, y compris ceux qui supposeraient une nouvelle intervention du législateur. Il y a la question de la vaccination obligatoire des soignants, que vous avez évoquée ; on peut aussi parler du recours au pass sanitaire, pour inciter encore plus de personnes à se faire vacciner ; et j'ai moi-même cité les questions de l'isolement au terme de la stratégie « tester,

pour éviter que les plus vulnérables à la maladie ne contractent le virus, parce que ce sont eux qui ont statistiquement la plus forte probabilité d'aller dans les services hospitaliers et de réanimation, qui sont, comme vous le savez, le goulet d'étranglement de cette épidémie.

Monsieur le Premier Ministre, les résultats sont tombés dimanche soir : votre majorité a subi un échec sans précédent ! Aucun président de région ou de département n'est issu des rangs de la majorité présidentielle ; vos ministres, et donc votre politique, ont été sèchement le secrétaire d'État chargé des retraites à 9,7 % dans les Hauts-de-France ; le garde des sceaux à 8,67 % dans le Pas-de-Calais ; la ministre de la transformation et de la fonction publiques à 11,21 % en Essonne, etc. Les déplacements très politiques et très médiatisés du Président de la République n'y ont rien changé : à Saint-Cirq-Lapopie, votre candidat a obtenu 3,7 %. Jamais le parti d'un Président de la République en exercice n'aura à ce point été rejeté par les électeurs ! Comment expliquez-vous, monsieur le Premier ministre, ces résultats ? expliquez-vous à la fois l'abstention record et la déroute des candidats appartenant à votre majorité ? Quelles conséquences allez-vous tirer de votre échec ? Allez-vous changer de politique ? Je suis un sénateur gaulliste, et vous êtes Premier ministre. Je respecte hautement votre fonction, mais vous devez incarner l'unité. J'aurais aimé échanger avec vous, voilà trois jours, lors de votre visite en Eure-et-Loir. Or vous avez snobé les sénateurs en oubliant de les convier à un logique accueil républicain. Ce jour-là, vous avez préféré la division à l'unité.

S'il est un enseignement national que nous pouvons toutes et tous tirer, et vous y avez fait référence, c'est le niveau abyssal de l'abstention à l'occasion de ces élections. Jamais, à un scrutin,

l'épidémie, depuis plus d'un an, fait que, probablement, un certain nombre de Français avaient la tête ailleurs. À l'occasion des dernières municipales, on a aussi constaté une baisse de participation de 20 points par rapport aux municipales précédentes, un chiffre que l'on retrouve pour les régionales. Il y a aussi des raisons plus structurelles, qui tiennent à notre organisation territoriale.

de construire pour l'avenir et de s'implanter progressivement. En tout cas, nous aurons toutes et tous des réflexions à mener et des conséquences à tirer de cette très faible participation. Monsieur le Premier ministre, comme nous, vous voulez faire reculer l'abstention, alors cessez de fustiger les électeurs ! Cessez d'opposer « nouveau monde » et « ancien monde », de prêcher qu'il n'y a ni gauche ni droite ! Mettez fin à l'absence de clarté et de convictions ! Fixez un cap et tenez-le ! Enfin, vous de mépriser les élus issus du suffrage universel en privilégiant les commissions ou comités de citoyens tirés au sort. Ainsi, vous réduirez l'abstention ! Monsieur le Premier ministre, n'ayez pas peur d'écouter et de suivre les recommandations du Sénat, car, ici, il n'y a que des élus qui aiment la France.

Bien sûr, supprimer ces épreuves chronophages et complexes à organiser va libérer du temps pour les élèves et les enseignants, et répondre mieux aux attentes de travail régulier et continu. Pour autant, cette mesure est très loin d'être mineure : faire reposer le baccalauréat pour 40 % sur les notes du livret scolaire fait peser un risque non négligeable de rupture d'égalité devant ce diplôme.

Rappelons que ces fameuses notes sont aussi la base des choix pour Parcoursup. Rappelons enfin que la crise sanitaire, avec un baccalauréat reposant essentiellement sur le contrôle continu, a montré de très importantes disparités de notation, sources de conflits et de critiques. Il ne saurait donc être acceptable que cette mesure ajoute de l'inégalité là où, déjà, les déterminants géographiques et sociaux font peser un poids très lourd sur la réussite des élèves. Ce dernier sujet, qui est majeur, n'a d'ailleurs pas trouvé sa réponse dans la réforme mise en oeuvre. Ma question est donc simple, monsieur le ministre : alors que, à peine appliquée, vous faites déjà évoluer la réforme du baccalauréat, quel cadrage allez-vous proposer pour garantir une égalité réelle de notation pour les lycéens, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont scolarisés ? Comment, et par qui cela sera-t-il suivi,

; 40 % de contrôle continu pour favoriser le travail continu de l'élève en première et en terminale. Je le répète, cela ne change pas : ce qui change, c'est que, à l'intérieur des 40 %, au lieu d'avoir les épreuves communes que nous avions installées voilà deux ans, il y a tout simplement le contrôle continu à l'échelle de l'établissement.

Monsieur le ministre, vous comprendrez que nous soyons inquiets, et le flou de votre réponse aggrave cette inquiétude. Où en est la promesse d'égalité républicaine, qui justifiait cette réforme, quand la première mesure d'ajustement est, au contraire, potentiellement source de plus d'inégalité ? Où en est-on, monsieur le ministre, des mesures visant à ce que les jeunes des quartiers et des territoires ruraux aient les mêmes chances que ceux des centres-villes, alors que l'ascenseur social est en panne ? Il faudra contrôler cette évaluation, et de très près

c'est au lendemain d'une bérézina électorale d'une ampleur inédite pour une majorité présidentielle que la réforme des retraites est de nouveau annoncée. L'âge de départ serait ainsi reporté à 64 ans, et cette mesure pourrait être adoptée en quelques lignes intégrées au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chaque parlementaire ici présent pourra apprécier la démarche pour le moins cavalière s'agissant d'un sujet aussi structurant et fondamental dans notre société. Certains ministres semblent craindre d'importants troubles sociaux, d'où les hésitations perceptibles ces derniers jours. Monsieur le Premier ministre, ma question est très simple, très claire : quelles sont exactement les intentions du Gouvernement sur ce projet de réforme des retraites ?

le Président de la République l'a dit, notre priorité absolue, aujourd'hui, c'est la sortie de la crise sanitaire, le rebond de notre économie et la création d'un maximum d'emplois. en sortie de crise, des questions qui se posaient sur notre système de retraite restent toujours d'actualité. Le rapport remis la semaine dernière par les économistes Jean Tirole et Olivier Blanchard conforte ce diagnostic. Il nous faut donc trouver les voies et moyens d'un système plus lisible, plus juste et plus soutenable. L'éclatement en quarante-deux régimes rend notre système de moins en moins adapté aux parcours professionnels de celles et ceux, toujours plus nombreux, qui changent de métier. Par ailleurs, on le sait, le système actuel pénalise les carrières hachées et les temps partiels souvent subis, situations vécues en particulier par les femmes. La question du financement des retraites demeure également fondamentale, comme le montrent les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites. Ainsi, il nous faudra travailler plus longtemps pour assurer le financement pérenne de notre système de retraite et la compétitivité de notre économie. Cela pose les questions du maintien dans l'emploi des seniors et, partant, de la formation tout au long de la vie, des reconversions lorsque c'est nécessaire et de la prévention de l'usure professionnelle. Ces sujets figurent à l'agenda social partagé avec les partenaires sociaux depuis juillet dernier. Dans ce contexte, le Président de la République a choisi d'entendre les Français, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les forces politiques. Je le redis, notre ambition reste la même

64 ans, ce sont deux années au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Nous vivons dans une société où les inégalités sont considérables. Nous constatons ainsi dix ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier de 59 ans et un cadre de 69 ans. Par ailleurs, 8 % des retraités survivent sous le seuil de pauvreté. Madame la ministre, la véritable question est celle-ci : quelle part de la richesse nationale sommes-nous prêts à consacrer au financement de notre système de retraite par répartition. C'est non pas une contrainte comptable et financière, mais un choix politique, un choix de société. Pour le financement, il conviendrait de remettre à plat la logique des allégements de cotisations sociales, par exemple. Il vous faudrait également élargir l'assiette des cotisations aux revenus financiers, qui se développent dans des proportions hallucinantes en dépit de la pandémie. Or, depuis l'instauration du prélèvement forfaitaire unique, ceux-ci ne sont plus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Madame la ministre, vous êtes face à un choix de société : un choix, vous dis-je

Ce lundi, les vingt-sept ministres européens de l'agriculture ont trouvé un accord sur la nouvelle politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027. Trois années de négociations ont été nécessaires pour aboutir à ce compromis et surmonter les points de divergence persistant entre les institutions européennes et les États membres. La nouvelle réforme de la PAC entrera en vigueur le 1 janvier 2023, après deux années de transition. Ce compromis était attendu à Bruxelles, à Paris, mais, surtout, par les premiers concernés sur nos territoires, à savoir nos agriculteurs. En juillet dernier, les chefs d'État européens s'étaient déjà accordés sur un budget renforcé pour la PAC. La France avait atteint son premier objectif en obtenant 62,4 milliards d'euros sur la période 2021-2027, soit 400 millions d'euros de plus qu'à l'occasion de la précédente programmation. L'aboutissement de cette réforme a nécessité d'âpres discussions au niveau européen, notamment sur le verdissement de notre agriculture, la simplification,

la création de valeur dans les exploitations agricoles sur nos territoires et la reconquête de notre souveraineté alimentaire au niveau national. Monsieur le ministre, ma question est simple : l'accord trouvé ce lundi conforte-t-il les choix de mise en oeuvre

effectivement, après trois années de négociations, nous sommes arrivés à un accord politique sur cette nouvelle politique agricole commune, voilà quelques heures, à Bruxelles, avec l'ensemble de mes homologues.

des financements assurés, une vision économique, environnementale et sociale affirmée : tel est le contenu de l'accord que nous avons conclu, et c'est un bon accord pour la France ! La parole La parole est à M. Patrick Kanner, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

et Républicain. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement et le Président de la République affrontent une séquence calamiteuse, marquée par un triple fiasco. Le fiasco de la propagande électorale : la commission d'enquête sénatoriale fera son travail. Le fiasco démocratique : avec 20 points de participation en moins par rapport aux élections de 2015, c'est une alerte majeure, dont nous devons collectivement tirer les conséquences. Le Président de la République, une grande légèreté, donne comme simple explication : « Les gens n'avaient pas du tout la tête à cela. » Quel manque de considération pour le travail des élus locaux et, surtout, quel mépris pour les citoyens ! Enfin, c'est un fiasco électoral pour La République En Marche, ce parti « virtuel » composé de « cliqueurs », comme le qualifie le président Patriat, et donc pour le Président de la République lui-même, qui était, malgré ses dénégations, la véritable tête de liste de ces élections. Je vous renvoie à son tour de France ou aux candidatures du tiers de ses ministres, avec le résultat que l'on connaît. Conséquence de la verticalité du pouvoir que vous avez installée depuis 2017, ce sont non seulement les élections territoriales que les Français ont boudées, mais, surtout, votre politique et l'action personnelle du chef de l'État. Pas du tout ! Alors, monsieur le Premier ministre, pour tirer les conclusions de ce triple fiasco, et plutôt que de relancer une réforme des retraites injuste et totalement décalée en cette période, je vous fais une proposition, qui, d'ailleurs, aurait le mérite de satisfaire un engagement présidentiel, une parole donnée en 2017 : débattez ! Débattez avec le Parlement en convoquant, dès juillet, le Congrès, sur le fondement de l'article 18 de la Constitution. Nous sommes les représentants de la Nation. Nous avons des choses à vous dire sur l'état de la France et sur votre bilan.

du Congrès qui aurait pu drainer davantage de nos concitoyens à ces élections, je vous laisse la responsabilité de cette appréciation Il est quand même curieux- ce n'est pourtant pas la première fois que je l'entends -que l'on nous reproche d'avoir voulu « nationaliser » ces élections,

les nationaliser que le Gouvernement de la République considère qu'il s'agit d'élections secondaires. Ce sont des élections extrêmement importantes pour la démocratie locale. Monsieur Kanner, je suis, comme vous,

-traiter la question des graves dysfonctionnements qui ont caractérisé l'acheminement des plis et de la propagande électorale,

toujours se renvoyer la balle, mais je crains que cela n'alimente encore davantage le désintérêt de nos concitoyens. Je vous le dis comme je le pense

dans vos fonctions ! Vous restez donc notre interlocuteur. Je vous ai fait une proposition ; je n'ai pas entendu un mot de vous à son propos. J'aimerais simplement que vous rappeliez à M. le Président de la République qu'il avait pris un engagement en 2017 : réunir le Congrès une fois par an pour faire le bilan de la situation de la France. Je vous réitère cette demande,

Les effets médicaux et psychosociaux de la crise du covid-19 affectent durablement notre jeunesse, et ce dès l'enfance. Même si nous saluons le maintien maximal de la présence à l'école, des séquelles Le suivi en médecine scolaire a été perturbé. La situation d'indigence de la médecine scolaire dans notre pays doit nous alerter davantage encore : un seul médecin pour 12 000 élèves Parallèlement, la protection maternelle et infantile (PMI) est confrontée aux mêmes problèmes de recrutement. Pourtant, la santé de nos enfants- leur état de bien-être physique, mental et social -bénéficierait d'une mutualisation et d'une complémentarité des services de médecine scolaire avec la PMI et les services sociaux des départements. Alors que nous envisageons les mesures sanitaires à prendre pour la prochaine alors que les départements renouvellent leurs exécutifs, l'organisation de leurs missions et de leurs services, n'avons-nous pas une formidable occasion de réunir ces services pour plus d'efficacité et d'exhaustivité dans ce contexte de pénurie de professionnels de santé, professionnels qu'il convient de ménager en les délestant des problèmes sociaux intercurrents ? Il existe une véritable logique de dépistage et d'accompagnement des enfants de la naissance à la fin de leur scolarité. Le 17 décembre dernier,

trouve effectivement la création d'un service de santé de l'enfant qui réunirait les moyens et les missions de la PMI et de la médecine scolaire. Cette proposition est d'ailleurs soutenue par l'Assemblée des départements de France.

Je vous propose donc que nous continuions d'y travailler ensemble. Territoires. Madame la ministre, y aura-t-il un avenir, dans notre pays, pour l'industrie automobile ? Avec autant de destructions d'emplois depuis vingt ans, la question est sérieuse. Dans ma région, je suis particulièrement sollicité

répondent ensemble la CFDT Métallurgie et la Fondation Nicolas Hulot, qui viennent de publier un rapport essentiel sur ce sujet. C'est du sérieux ! Cette contribution majeure au débat indique un chemin viable sur notre sol national pour une industrie automobile combinant emploi et écologie. Quatre scénarios sont comparés : il en ressort que seule la transition écologique accélérée du secteur automobile permettra de maintenir durablement en France la production et le savoir-faire. Ils en appellent pour cela à des états généraux de l'automobile, afin que le dialogue social, industriel et sociétal puisse converger sur les conditions d'un scénario positif pour l'emploi et le climat : en clair, une stratégie industrielle partagée. Madame la ministre, j'ai donc deux questions à vous poser. Le Gouvernement est-il résolu à engager cette démarche ?

nos paroles, nos plaidoyers pour cette industrie, en conformité avec nos actes, avec les décisions que nous prenons à tous les niveaux pour faciliter l'implantation de nouveaux sites industriels et favoriser l'emploi industriel. C'est de cela aussi qu'il est question

de la batterie électrique.

toute orientation objective ? Estimez-vous de bonne conduite que des élèves candidats aux concours des grandes écoles puissent désormais bénéficier, par avance, de points supplémentaires sur des critères qui s'apparentent essentiellement à de la discrimination positive ? Croyez-vous qu'au concours de l'École polytechnique les mathématiques et la physique ne soient plus suffisantes pour choisir les meilleurs ? Ne craignez-vous pas, en définitive, que ces évolutions auxquelles tiennent tant certaines élites qui ont pu y échapper se fassent au détriment du rayonnement des formations supérieures et, surtout, de l'équité que l'on doit aux élèves ?

qui promeut le mérite. Oui, aujourd'hui, nous constatons plus de mobilité sociale et une meilleure représentation des boursiers dans toutes les formations, y compris les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est le résultat concret de la lutte contre l'autocensure que nous ne cessons de mener. Dans le même temps, la réussite à l'université a progressé.

Je vous rappelle d'ailleurs que les concours d'accès aux grandes écoles ont tous été préservés et maintenus l'an dernier, malgré la crise sanitaire et grâce au travail mené par le Gouvernement, en lien avec les écoles. Maintenant, regardons les chiffres,

monsieur les ministres, je n'aurais jamais cru que, sous votre magistère collectif, on s'éloignerait davantage encore de la promesse républicaine qui a vu Charles Péguy, le fils d'une rempailleuse de chaises, devenir normalien, ou Albert Camus, le fils d'une femme de ménage, recevoir le prix Nobel de littérature, tout cela sans quotas Je n'aurais jamais cru que ce serait sous votre magistère que l'excellence et le mérite, mesurés par le travail, les connaissances et l'effort, seraient abaissés au rang d'incongruité ! J'avais pourtant sincèrement espéré que vous fermeriez la porte à cette fascination pour les délires wokistes venus d'outre-Atlantique, pour lesquels s'entichent ceux qui sont si prompts à passer par-dessus bord tout ce qui a forgé notre modèle républicain. J'espérais que vous auriez fait vôtre cette belle citation de Philippe Nemo Ce n'est pas en faisant injure aux valeurs de raison, de science, d'intelligence et de travail qu'on forme la jeunesse d'un pays. » Madame, monsieur les ministres, c'est bien sous votre magistère, hélas, qu'à bas bruit nous tournons le dos à la méritocratie républicaine La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre assemblée a adopté hier le projet de loi Climat. Notre groupe politique a voté contre ce projet en l'état, considérant qu'il n'était pas à la hauteur de l'enjeu climatique. Nous savons tous ici que les forêts, en tant que puits de carbone, sont l'un des leviers de la transition écologique et de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, qui implique une politique forestière ambitieuse, rationnelle et durable. Pourtant, depuis des années, l'instrument national qui est chargé d'assurer cette gestion et cet entretien, l'Office national des forêts (ONF), ne bénéficie pas d'une attention suffisante des pouvoirs publics. Il est en déficit structurel, sans véritable modèle économique permettant de lui assurer stabilité et développement. Un nouveau cadre contractuel avec l'État est en discussion. Toutefois, comme nous l'avons évoqué lors des débats sur le projet de loi Climat, ce que nous en savons nous inquiète particulièrement. citer la réduction envisagée du personnel, alors que l'ONF a déjà perdu 40 % de ses effectifs en vingt ans ; cette situation suscite une très forte inquiétude des personnels de cet office, qui ne voient pas comment ils pourront, demain, faire plus avec moins de moyens. Ajoutons-y le recours systématique et grandissant aux collectivités territoriales pour contribuer au budget de l'ONF. Dans le projet gouvernemental, l'augmentation de la contribution des communes s'élèverait à près de 30 millions d'euros pour les budgets de 2023 à 2025. Nos communes forestières s'insurgent contre cette nouvelle ponction, dont nous savons par ailleurs qu'elle ne suffira pas à recréer l'équilibre budgétaire et la stabilité durable de l'ONF. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de travailler sincèrement à un plan de renforcement des moyens de l'ONF qui permette de relever véritablement le défi du réchauffement climatique, en veillant particulièrement au personnel de cet office et sans grever davantage encore le budget des communes

Comme chaque année depuis trois ans, la ville de Grenoble est en pointe sur le sujet ! Cette polémique est parfaitement orchestrée autour de trois acteurs. Tout d'abord, on trouve un maire écologiste, candidat déclaré à l'élection présidentielle ; pour séduire un électorat, il entretient la polémique quant à sa position sur le sujet et renvoie la responsabilité à votre gouvernement. Ensuite, il y a une association militante, qui a d'ores et déjà annoncé mener des actions de désobéissance civile

Mme la ministre déléguée chargée de la citoyenneté affirmait quant à elle en mars dernier : « Nous faisons face à une petite minorité qui promeut un islam radical et rétrograde, notamment pour les femmes.

Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin d'entendre le Gouvernement clarifier sa position ; nous ne pouvons accepter de telles postures, qui sont un réel danger pour notre vie en société. Aussi, monsieur le Premier ministre, quelle est la position de votre gouvernement sur le port du burkini ? Quelle règle souhaitez-vous voir appliquer dans nos territoires ? Enfin, êtes-vous favorable à l'organisation d'un référendum local sur ce sujet ?

On demande aujourd'hui aux élus de petites communes rurales, souvent démunies en services, d'accueillir du public en toute sécurité, d'assumer les dégâts croissants que cause le gibier sur de jeunes plantations, d'approvisionner en priorité les entreprises françaises et les filières de construction, et de réguler les marchés par leur flux, quitte à reporter des ventes pourtant attendues, voire à perdre des recettes. Dans ce contexte de crise forestière et de guerre commerciale mondiale sur les matériaux, les communes forestières servent l'intérêt général sans recevoir, jusqu'à présent, aucune compensation financière.

Quelles suites allez-vous donc donner à ces mesures irréfléchies et à cette absence de plan d'avenir pour la forêt française ?

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour le groupe Les Républicains Madame la ministre, depuis des semaines, deux France s'affrontent : celle des Français qui aspirent à un retour à la normale, à l'allégement de toutes les restrictions, et celle des Français qui regardent l'avenir avec inquiétude, tant est grand le risque d'une reprise épidémique à la rentrée. je fais partie des Français inquiets. De nombreux pays freinent leur déconfinement, alors qu'en France, dès aujourd'hui, il n'y a quasi plus de restrictions, que la vaccination stagne, que des clusters apparaissent et que débutent les grandes migrations estivales.

que l'on pouvait y échapper. La France serait-elle la seule à y échapper ? Le Gouvernement n'a ni prévu ni anticipé l'épisode de relâchement de l'été dernier, encore moins l'invasion rapide du variant anglais cet hiver. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'annoncer que vous aviez anticipé en créant une consultation. Allez-vous agir immédiatement et pendant l'été ? La menace d'une vaccination obligatoire des soignants au mois de septembre prochain n'est pas suffisante et la rentrée universitaire et scolaire n'est jamais évoquée. Ma question est simple : cette année, avez-vous au moins un plan dans les cartons ou allez-vous encore naviguer à vue ?

Le taux d'incidence est de 18,5 pour 100 000, soit plus de vingt fois inférieur à celui qui a justifié le renforcement des mesures sanitaires qui prennent donc fin ce jour. Dans le même temps, le taux de positivité des tests est inférieur à 1 % et le nombre d'hospitalisations pour cause de covid-19 connaît une baisse considérable, puisque nous sommes passés sous la barre des 8 700 lits occupés, dont 1 260 en réanimation. Si cette situation a été rendue possible, c'est pour deux raisons. D'une part, les Français ont été à la hauteur, ont respecté les consignes sanitaires, car celles-ci étaient proportionnées et ont porté leurs fruits.

un Français sur deux a désormais au moins reçu une dose de vaccin et 22 millions de Français bénéficient d'un schéma complet. Notre ligne de conduite consistant à « tester, alerter, protéger » a toujours été accompagnée de la réponse la plus fine possible à une situation donnée pour préserver notre système de santé. Néanmoins, certains variants, vous l'avez indiqué, madame la sénatrice, gagnent du terrain dans le monde entier et arrivent dans notre pays : ils représentent désormais 20 % des contaminations, tout en étant de 60 % à 90 % plus transmissibles. Bien sûr, nous tâchons de circonscrire le plus possible cette situation en accompagnant au cas par cas dans les territoires. Par exemple, dans le département des Landes, un plan d'action renforcé est lancé avec une augmentation du nombre de doses de vaccins disponibles, un renforcement de la démarche d'« aller vers », le, mais également, quand cela est nécessaire, des mesures de freinage. De la même façon, le déploiement du pass sanitaire est un outil de protection renforcée et nous allons le développer. La réponse de l'État est là, mais le civisme de chacun d'entre nous est la seule assurance d'éviter une quatrième vague. Je le rappelle, les vaccins disponibles protègent à 90 % des formes graves après une couverture vaccinale complète. vous n'annoncez absolument rien de nouveau ! Je ne conteste pas que la situation soit bonne, mais je vous demande ce qui est prévu pour éviter une quatrième vague. L'Académie de médecine a proposé de rendre les tests de confort payants

les non-vaccinés seront confinés ou confinera-t-on tout le monde ? Les Français sont inquiets et on aimerait avoir des réponses, des réponses rapides et des réponses d'anticipation. Ce n'est pas le cas cet après-midi.

Les Français de l'étranger sont, depuis le début de la campagne vaccinale, incités par votre gouvernement à se faire vacciner dans leur pays de résidence. Selon les pays, les vaccins diffèrent et tous ne sont pas reconnus par la France. Ainsi, un Français vacciné avec Sinovac ou Spoutnik sera considéré comme « non vacciné » s'il souhaite rentrer en France : il sera alors soumis à son arrivée à un auto-isolement ou à une quarantaine surveillée. Pourtant, une partie significative de ces vaccins sont obtenus par l'initiative Covax, qui a pour finalité de distribuer des vaccins dans les pays ne disposant pas de la capacité d'en acquérir.

De surcroît, ceux qui auraient été vaccinés à l'étranger avec un vaccin reconnu en France peuvent voir leur certificat de vaccination étranger reconnu « au niveau des frontières pour entrer en France », mais celui-ci ne permettra pas pour autant l'accès aux événements soumis au pass sanitaire. Un test récent PCR ou antigénique négatif devra alors être présenté ! Rien ne justifie cela : soit l'attestation vaccinale étrangère avec un vaccin reconnu en France est valable, soit elle ne l'est pas ! Enfin, si le Gouvernement a annoncé que la France organisait la vaccination à l'attention des Français de l'étranger dans pays, aucune liste n'a été communiquée à ce jour ni aucune stratégie globale présentée. Nos compatriotes nous sollicitent chaque jour afin d'obtenir des informations concernant la stratégie vaccinale de la France, tant les incertitudes et difficultés pratiques sont présentes. Ces sujets sont aussi essentiels pour les touristes appelés à visiter la France au cours de l'été. Quelles sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à faire preuve d'une telle incohérence concernant les certificats vaccinaux étrangers ? Quand cessera l'hypocrisie consistant à participer à l'initiative Covax pour la distribution de vaccins, alors que de nombreux vaccins administrés par cette voie ne sont pas reconnus en France ?

et pour en faire un bien public mondial. La solidarité vaccinale, dont le dispositif Covax est la meilleure incarnation, est un impératif moral, mais aussi la seule façon de mettre fin ensemble à la pandémie. La France est aux côtés des siens, où qu'ils soient dans le monde. Elle est le seul pays à avoir lancé la vaccination de ses communautés à l'étranger. Certains de nos partenaires ont des plans de vaccination, mais uniquement pour leurs agents publics expatriés. Dès le mois de décembre des travaux ont été lancés en ce sens, avant même que la vaccination ne débute sur le territoire national. De premières doses ont été envoyées au début du mois de mai dernier en Inde, à Madagascar. Désormais, c'est dans plus de que des doses ont été envoyées ou sont en cours d'envoi. Des envois supplémentaires sont à l'étude. Cette vaccination s'appuie sur le réseau diplomatique et consulaire, avec l'appui des autorités sanitaires partenaires. Ce sont des opérations lourdes, qui demandent l'accord des pays dans lesquels elles sont réalisées. Les autorisations ne sont parfois pas encore données, nous y travaillons. Avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, nous allons simplifier et amplifier nos efforts pour nous inscrire dans une géographie plus vaste et dans un temps long. Par ailleurs, nos compatriotes de l'étranger peuvent tous se faire vacciner gratuitement sur le territoire national, les délais d'injection entre deux doses étant réduits à vingt et un jours. Pour ceux qui reviennent d'un pays en liste rouge, soumis à une quarantaine administrative et non à un isolement, il est possible de sortir quelques heures par jour pour des motifs essentiels, essentiels, dont la vaccination fait partie. Enfin, pour ce qui est des types de vaccins reconnus, seuls les vaccins homologués par l'Agence européenne des médicaments sont employés, car notre unique préoccupation est l'efficacité vaccinale. L'homologation du vaccin AstraZeneca dans sa version Covishield est à l'étude par l'Agence européenne des médicaments. Elle interviendra dans les meilleurs délais. Pour ce qui est des frontières, nous sommes très attentifs à la situation épidémique mondiale. Le dispositif-cadre de la coordination européenne, dont la France est motrice, s'adapte pour assurer la meilleure protection des Français. La parole est à M. Vincent Segouin, pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Madame la ministre, les agents généraux d'assurances sont inquiets ! Comme vous le savez, le financement du régime de retraite des agents généraux d'assurances est fondé sur une cocontribution financière des agents généraux et des compagnies d'assurances. Ce cofinancement est la conséquence de l'interdépendance économique qui existe. Aussi, actuellement, un agent général doit partir à la retraite à 67 ans pour bénéficier il cotise sur son chiffre d'affaires, peu importe son bénéfice. Leur caisse de retraite est la seule qui agisse ainsi. Jusqu'à présent, la contribution des compagnies d'assurances a toujours été de 3 % du chiffre d'affaires. Le dernier accord arrive à échéance au 31 décembre 2021. Or il se trouve que les compagnies d'assurances ont décidé de se désengager totalement du financement du régime de retraite des agents généraux. Cette décision est incompréhensible au regard des bénéfices annuels publiés par ces mêmes compagnies. Ce désengagement total conduirait à une augmentation de 58 % des cotisations des actifs, à une baisse de 33 % des droits à retraite ou à l'épuisement de la caisse dans les deux ans.

l'Orne. Depuis 1952, des accords conventionnels successifs prévoient la prise en charge par les compagnies d'assurances d'une partie des cotisations des agents généraux d'assurances à leur régime de retraite complémentaire. Cela représente actuellement environ 90 millions d'euros par an, soit plus du tiers des ressources du régime. L'accord aujourd'hui en vigueur expire à la fin de l'année. Des négociations sont donc en cours entre les organisations représentatives des compagnies d'assurances et des agents généraux. Il semble, comme vous l'avez indiqué, que les compagnies d'assurances aient fait savoir qu'elles souhaitaient se retirer d'une partie de cette prise en charge des cotisations, ce qui compromettrait encore plus l'équilibre financier déjà précaire malgré les réserves importantes- de l'ordre de 1,3 milliard d'euros en 2019 -, le régime est structurellement en déséquilibre technique. Très respectueux des dispositifs conventionnels, l'État n'a pas vocation à se substituer à l'une des parties ni à empêcher que ces relations évoluent. Pour autant, un désengagement brutal des compagnies d'assurances mettrait en réelle difficulté le régime de la caisse Celui-ci a en effet une obligation réglementaire de disposer d'une visibilité à quarante si l'État n'entend pas se substituer à ce dispositif conventionnel, il est attentif aux négociations en cours et à leurs conséquences sur le régime des agents d'assurances. Le Gouvernement sera particulièrement vigilant à ce que l'accord qui sera trouvé entre les parties garantisse l'équilibre de long terme du régime, comme le prévoit la réglementation, et également les droits des affiliés.

et de l'alimentation. Les agriculteurs sont inquiets de la renégociation des contrats d'achat d'électricité photovoltaïque. Contre l'avis du Sénat, le Gouvernement a voulu réviser les tarifs d'achat de l'énergie produite par les installations photovoltaïques. Le Sénat avait pourtant mis en garde sur le signal désastreux que cette négation des engagements de l'État enverrait à l'ensemble de la filière des énergies renouvelables, mais également sur la menace qu'elle ferait peser sur les exploitations agricoles. Le 2 juin dernier, le Gouvernement a rendu publics les nouveaux tarifs en se fondant sur les calculs de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Alors que le Gouvernement promettait une baisse moyenne de 55 %, de nombreux agriculteurs bailleurs de toitures pourraient connaître des baisses allant jusqu'à 95 % du prix Cette révision avait pourtant été validée par le Conseil constitutionnel à la condition qu'elle n'affecte pas la viabilité économique des structures de production et assure une rentabilité raisonnable à ces nombreux agriculteurs qui, pendant des années, ont contribué au développement des énergies solaires. L'État manquerait-il aujourd'hui à sa parole ? Cette double peine est infligée aux agriculteurs sur la base de calculs théoriques de la CRE, déconnectés du terrain et des réalités économiques. Elle aurait des conséquences financières désastreuses pour les porteurs de projets et les bailleurs. Avec un prix de revente qui pourrait être divisé par au moins dix selon les syndicats agricoles, comment feraient les agriculteurs pour rembourser leurs emprunts, payer les charges ou assurer la rentabilité des installations ? Monsieur le ministre, pouvez-vous garantir que le Gouvernement tiendra ses engagements, respectera la volonté du législateur et assurera une sécurité juridique et financière aux agriculteurs qui se sont engagés de bonne foi pour l'environnement ?

aux zones non interconnectées et aux acteurs agricoles et nous prévoyons une clause de sauvegarde qui permette aux exploitants de demander une analyse individuelle de leur situation par la Commission de régulation de l'énergie, afin de pouvoir conserver des conditions de rémunération qui soient satisfaisantes. je rappelle que cette révision s'applique aux contrats qui relèvent d'installations dont la puissance est supérieure à 250 kilowatts-crête, soit plus de 3 000 mètres carrés de panneaux solaires- je vous laisse imaginer l'importance de ces exploitations qui exclut de ce dispositif les particuliers et la plus grande majorité des agriculteurs. Cette mesure est justifiée d'un point de vue budgétaire. Elle ne remet en aucun cas en cause l'objectif gouvernemental d'un soutien massif au développement des énergies renouvelables, comme en témoignent les 110 milliards d'euros d'engagements sur les vingt ans à venir, l'augmentation de 25 % du soutien financier aux énergies renouvelables entre 2020 et 2021 et des appels d'offres d'ores et déjà prévus pour plus de 10 gigawatts d'installations photovoltaïques au cours des cinq prochaines années. Ce sont autant d'installations qui peuvent constituer utilement un complément de revenu agricole agricole et qui participent à la transition énergétique française. La parole à quinze heures. J'informe le Sénat que, conformément à l'article 8 du règlement, les listes des candidats remises par les groupes politiques pour participer à la mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences ont été publiées.